Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, c’est avec émotion et tristesse, particulièrement pour ceux qui l’ont connu, que nous avons appris hier la mort de Jacques Valade.

adjoint au maire de Bordeaux en 1971, puis premier adjoint en 1977. En 1973, il fait son entrée au conseil général de la Gironde, dont il est élu président. prendra activement part à la campagne de Jacques Chaban-Delmas pour l’élection présidentielle de 1974, campagne qui le marqua profondément. Il devient sénateur le 28 septembre 1980. Il rejoint alors le groupe du Rassemblement pour la République (RPR) au Sénat et intègre la commission des affaires économiques et du plan. Il est alors désigné par son groupe pour le suivi de l’aménagement du territoire. Il est ainsi au cœur des grandes lois de décentralisation portées par Gaston Defferre en 1982. Il rappelle alors combien la Haute Assemblée porte la voix des collectivités territoriales. Il aura l’occasion de mettre à profit ses compétences universitaires et scientifiques en 1987 lorsque Jacques Chirac lui demande de succéder à Alain Devaquet en tant que ministre délégué, chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur auprès de René Monory.

Il s’impliquera alors dans la création de Public Sénat. En 2001, il devient président de la commission des affaires culturelles. Il sera rapporteur du projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sujet qui demeure d’actualité. Nous garderons de Jacques Valade le souvenir d’un parlementaire très impliqué dans ses missions de législation et de contrôle, d’un élu profondément attaché à la ville de Bordeaux et à la Gironde, mais aussi d’un scientifique exigeant, doté d’une culture très étendue et d’une vive curiosité intellectuelle. Au nom du Sénat,

Mes chers collègues, c’est aussi avec émotion que nous avons appris hier le décès de Jean-Pierre Elkabbach.

Il devint président de Public Sénat en décembre 1999, fonction qu’il assuma pendant dix ans, s’attachant à mettre en valeur les travaux et l’image de notre assemblée.

Le passionné de littérature qu’il était anima avec talent l’émission. Au fond, il a su rendre plus accessibles nos institutions

L’ordre du jour appelle la désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat et la proclamation de la constitution du bureau définitif. Conformément à l’article 2 du règlement, la liste des candidats à chacune de ces fonctions a été publiée à douze heures trente. Cette liste n’a fait l’objet d’aucune opposition pendant le délai réglementaire.

Conformément à l’accord intervenu entre les présidents de groupes politiques, Mme Céline Brulin remplacera M. Joël Guerriau en qualité de secrétaire du Sénat à compter du 1 avril

Je déclare le bureau du Sénat constitué. Communication en sera donnée à M. le Président de la République, à Mme la Première ministre et à Mme la présidente de l’Assemblée nationale.